La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation et de programmation renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Votre texte a pour objet louable de mieux lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Nous partageons, en effet, le constat que les violences sexuelles et sexistes sont un fléau, qu'il faut dénoncer et combattre. L'actualité des derniers jours le démontre encore. Je souhaite revenir sur l'historique de notre accord aujourd'hui. Car bien des revirements ont finalement débouché sur un texte utile, qui porte la marque du travail approfondi effectué Concernant la répression des viols commis à l'encontre des mineurs, rappelons que la proposition initiale du Gouvernement était inopérante, car contraire aux principes fondamentaux qui régissent notre droit. Elle instaurait une présomption irréfragable de culpabilité pour l'adulte qui aurait commis un acte sexuel avec pénétration sur un mineur. C'était donc une responsabilité automatique que le Conseil constitutionnel n'aurait pas manqué de censurer.

nécessaire à la qualification de viol, soit caractérisée par le simple abus qui a été fait de la vulnérabilité de la victime. Il s'agissait là d'une mesure incitative pour le magistrat, déjà utilisée d'ailleurs par celui-ci. Vous proposiez également de créer une circonstance aggravante au délit d'atteinte sexuelle qui risquait de multiplier les correctionnalisations, ce que les associations ont, à juste titre, pointé du doigt. Cette proposition, avouons-le, n'avait d'autre objectif que de répondre à des impératifs politiques, voire médiatiques. Afficher un seuil d'âge aurait été sans conséquence sur la réalité de la protection de l'ensemble des mineurs. Le Sénat a choisi d'aller plus loin, en protégeant tous les mineurs victimes de viols, pas seulement ceux de moins de quinze ans, comme vous le proposiez, madame la secrétaire d'État, et pas uniquement ceux de moins de treize ans, comme l'a proposé, ensuite, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes du Sénat.

Cette solution de compromis, que certains d'entre vous trouveront peut-être timorée, mais que nous estimons conforme à notre État de droit, porte sur la caractérisation de la contrainte ou de la surprise pour les faits d'agression sexuelle commis sur mineurs. Il était, selon moi, essentiel de mieux définir les circonstances permettant au juge de retenir l'existence d'une contrainte ou d'une surprise, en prenant en compte la différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur des faits, ainsi que l'a toujours souhaité le Sénat, mais aussi « l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire » dans le cas spécifique des mineurs de moins de quinze ans, comme l'avait proposé l'Assemblée nationale. Il s'agit, vous l'aurez compris, mes chers collègues, d'un « dispositif à deux étages », comme l'a défini le président Philippe Bas, qui concernera tous les mineurs et s'appliquera aux agressions sexuelles comme aux viols. Je manquerais à mes devoirs si je ne mentionnais pas non plus les importantes évolutions adoptées par le Sénat. Je pense à la modification de la définition du délit de non-dénonciation de mauvais traitements, afin d'en faire un délit continu, mais aussi à la suppression de l'aggravation des peines en cas d'atteinte sexuelle avec acte de pénétration, ainsi qu'aux garanties apportées à la question subsidiaire systématique, sans oublier la définition du délit et des circonstances aggravantes en cas d'administration d'une substance visant à altérer le discernement d'une victime d'agression sexuelle. à l'aggravation des peines prévues pour toutes les agressions sexuelles lorsqu'elles sont commises sur une personne vulnérable en raison de sa situation économique et en cas d'agression sexuelle autre que le viol lorsque celle-ci a entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, ou encore à l'enrichissement des circonstances aggravantes des violences commises en présence d'un mineur et à la création d'un nouveau délit d'atteinte à la vie privée afin de réprimer « le fait d'user de tout moyen afin d'apercevoir les parties intimes d'une personne Plusieurs articles reprennent également la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles que nous avions adoptée le 28 mars dernier je songe aux dispositions concernant le délai de prescription des viols commis à l'encontre des mineurs, la répression du délit de non-assistance à personne en danger, ou encore l'extension de la surqualification pénale d'inceste. J'ai bien conscience que le travail n'est pas fini, et je suis déterminée à rester attentive et mobilisée. Nous devons convaincre, encore, que le sujet mérite un large consensus autour de mesures fortes et toujours plus efficaces visant à lutter contre toute forme d'agression sexuelle, en particulier celles qui de mineurs. Il est de notre responsabilité de protéger les enfants des prédateurs et des outils de communication qui peuvent les mettre en danger. C'est un enjeu crucial pour aujourd'hui et pour demain. Nous avons aussi l'obligation morale de nous occuper des plus faibles et des plus démunis. C'est même le ciment de notre vouloir-vivre ensemble. C'est une chance qu'il ne faut pas gâcher.

Madame la présidente, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le 25 novembre dernier, le Président de la République déclarait l'égalité entre les femmes et les hommes grande cause nationale de son quinquennat. Moins d'un an après, c'est un plaisir et un honneur d'être aujourd'hui devant vous pour conclure ensemble l'élaboration du projet de loi constituant l'une des pierres angulaires de cette démarche. La promesse faite à l'occasion de la dernière Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est tenue, et nous pouvons activement nous en féliciter. Le texte que vous vous apprêtez à voter en lecture définitive est le fruit d'un long travail, engagé depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, bien avant l'élection présidentielle. Une fois adopté, le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes sera ainsi la première grande loi citoyenne du quinquennat, grâce à la mobilisation des 55 000 participantes et participants au tour de France de l'égalité femmes-hommes, ce qui en fait la plus grande consultation gouvernementale jamais organisée. Mesdames, messieurs les sénateurs, beaucoup d'entre vous y ont largement contribué, et je veux vous en remercier. Lors de ces rencontres, partout en France, nos concitoyennes et nos concitoyens nous ont dit l'urgence d'agir pour faire reculer les violences subies quotidiennement par des millions de femmes dans pays. Ces échanges ont montré la nécessité de répondre à un triple objectif : mieux prévenir les violences, mieux accompagner les victimes, mieux sanctionner les agresseurs.

L'allongement à trente ans du délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur mineurs permettra une meilleure prise en compte des phénomènes d'amnésie traumatique et de la difficulté des victimes à parler des violences subies, particulièrement dans l'enfance. La caractérisation de la contrainte facilitée pour les agressions sexuelles et les viols commis sur des mineurs de moins de quinze ans est tout aussi importante. Affirmer qu'un mineur, en dessous d'un certain âge, n'est pas consentant à un acte sexuel avec un majeur constitue, à nos yeux, un véritable enjeu de civilisation. Cet objectif se trouve aujourd'hui renforcé par la disposition soutenue par votre assemblée, qui permettra de mieux prendre en compte également la différence d'âge entre la victime et l'agresseur, pour protéger l'ensemble des mineurs et mieux condamner les auteurs des violences qui sont infligées

les sénateurs, nous en avons eu une illustration récente dans l'actualité, puisque, la semaine dernière, une jeune femme a eu à subir ce phénomène de harcèlement de rue, qui s'est même poursuivi par des violences et une agression.

française, la liberté des femmes d'aller et venir comme bon leur semble et l'égalité entre les femmes et les hommes face à la question de l'occupation de l'espace public.

ces violences. Ces faits ont également permis à chacune et à chacun de se rendre compte de la réalité du harcèlement de rue que les femmes subissent depuis des générations.

Aujourd'hui, nous refusons cette fatalité et nous posons, avec le présent texte, un interdit social clair face au harcèlement quotidien que vit encore un trop grand nombre Au-delà de ces avancées majeures, le Gouvernement a souhaité réaffirmer sa volonté d'adapter l'arsenal répressif aux nouvelles formes de violences sexistes et sexuelles. Je pense notamment à l'inscription dans la loi de l'interdiction d'utiliser une substance, drogue du viol notamment, visant à altérer le discernement et de l'interdiction de ce que l'on a appelé le, en d'autres termes le voyeurisme, dont sont victimes de trop nombreuses femmes.

tant que la société tolérera que s'exercent de manière aussi massive des violences à l'encontre de toute une partie de la population, c'est-à-dire des femmes. Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi dont nous avons débattu, amélioré par les deux chambres, et adopté en commission mixte paritaire, est, je le crois, équilibré et assurément bien plus protecteur que le droit actuel. Je sais que toutes et tous vous partagez cette ambition, et je veux saluer l'engagement constant des deux chambres sur cette question, comme le montrent les travaux qui ont été conduits au sein des commissions des lois, mais aussi des délégations aux droits des femmes. Je crois que les enjeux portés par les textes amènent à construire des convergences. C'est ainsi que la commission mixte paritaire réunie la semaine dernière a permis d'établir un consensus là où certains auraient voulu créer des clivages. Je tiens donc à vous en remercier. Face à l'importance de l'enjeu, vous avez su trouver un terrain d'entente pour faire en sorte que le présent projet de loi, une fois adopté et promulgué, permette de mieux condamner les auteurs de violences et de mieux protéger les victimes. Vous n'avez eu que cet objectif en tête, et de cela je vous en sais Je suis ravie de constater que la sagesse et l'esprit de responsabilité l'ont emporté sur des positions partisanes. Vous avez su montrer que, au-delà des oppositions, les parlementaires travaillent ensemble, toujours avec le soutien du Gouvernement, et sont résolument mobilisés dans la lutte contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles. Certains nous avaient annoncé une loi clivante ; c'est, au contraire, une loi consensuelle qui sera votée aujourd'hui. Elle n'en est pas moins forte et ambitieuse. Le travail réalisé a été rendu possible uniquement parce que, indépendamment de la commission mixte paritaire conclusive, les parlementaires se sont saisis de ce texte et l'ont considérablement enrichi par de nombreuses contributions pour renforcer l'arsenal protecteur que nous sommes en train de construire ensemble.

engagé par le Président de la République : atteindre enfin l'égalité entre les femmes et les hommes, avec l'appui, je n'en doute pas, de l'ensemble des parlementaires. de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes vient aujourd'hui compléter l'édifice que nous sommes en train de bâtir pour changer le quotidien de toutes et tous. D'ores et déjà, les mesures que nous prenons contre ces violences permettent de mieux accompagner les victimes. Ainsi, dès la rentrée, nous mettrons en place des contrats locaux de lutte contre les violences, notamment intrafamiliales, qui assureront un meilleur repérage des victimes par un travail en réseau des professionnels de santé, de la justice, des forces de l'ordre et du tissu associatif. Le ministère de l'intérieur ouvrira en septembre prochain une plateforme de signalement, gérée par des policiers spécifiquement formés par la mission interministérielle pour la protection des femmes, pour informer et orienter les victimes de violences sexistes et sexuelles. J'ajoute que dix centres de prise en charge des psycho-traumatismes seront ouverts dans les territoires d'ici à la fin de l'année. Enfin, la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail est également une priorité. J'en veux pour preuve les dispositions du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui renforcent considérablement les moyens et les résultats exigés en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, ou l'appel à projets que nous avons lancé, pour un montant d'un million d'euros, afin d'épauler des initiatives soutenues par des organisations, des syndicats ou des associations. Vous le constatez, la politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est un ensemble : la loi n'est qu'un pilier parmi d'autres, indispensable, mais pas exclusif. La question de l'égalité est en jeu, partout, tout le temps, dans toutes les sphères de la société, et s'inscrit dans le plan global défendu par le Gouvernement. La rentrée sera l'occasion de faire de nouvelles annonces fortes, qui viendront compléter ce dispositif. Vous le savez, nous portons une attention toute particulière aux plus jeunes, comme le montre le travail que mon collègue ministre de l'éducation nationale et moi-même avons engagé, pour les sensibiliser, dès le plus jeune âge, pour mieux protéger les enfants en leur inculquant notamment le respect d'autrui, le respect de son corps, la notion de consentement. Ainsi, un référent égalité sera nommé dans chaque établissement scolaire, afin d'accompagner les élèves. Par ailleurs, les séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, prévues depuis la loi de 2001, seront obligatoires sur tout le territoire. Enfin, la mallette des parents intégrera des outils relatifs à la lutte contre l'exposition précoce à la pornographie, notamment. Dans la continuité, nous lancerons une grande campagne de communication à partir de la rentrée, avec des spots diffusés à la télévision, à destination des témoins.

Quand un voisin est en train de frapper son épouse, chez lui, dans son appartement, à l'abri derrière ses murs, ce n'est pas une affaire privée, c'est une question de de société, et il faut le dénoncer. Nous devons arriver à construire cette société de la vigilance, que le Président de la République a appelée de ses voeux quand il a lancé la grande cause nationale du quinquennat. Lorsqu'une femme est suivie, invectivée, entravée dans sa liberté, menacée dans la rue, dans l'espace public, il faut que les témoins interviennent. Quand on est témoin d'agressions sexuelles, de viols, d'agressions physiques, d'agressions sexistes, d'injures publiques envers les femmes, il faut aller déposer

Enfin, la question de l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, autre enjeu majeur, viendra s'adosser à la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui reste bien évidemment une priorité. Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement oeuvre à renforcer la protection des victimes, à mieux sanctionner les agresseurs. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles, qui ont trop souvent été tues ou « invisibilisées », est l'engagement du Président de la République que l'action de l'ensemble du Gouvernement traduit en actes, et que votre assemblée inscrit aujourd'hui dans la loi. Je connais votre engagement, sur l'ensemble de ces travées, en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je ne doute pas de votre implication. Je crois que, partout dans vos territoires, vous êtes les véritables garants, en tant qu'élus de la République, de cette égalité. J'espère que vous

de loi aborde un enjeu profondément humain : le respect de l'intégrité et de la dignité de chacun, des femmes et plus particulièrement des enfants. Le constat est partagé par tous : il est nécessaire de renforcer la protection des mineurs contre les infractions sexuelles et de réprimer le harcèlement de rue. L'actualité nous le rappelle régulièrement. Il y a eu l'affaire de Pontoise, ou encore l'agression dont a été victime Mme Marie Laguerre vendredi dernier : chaque jour charrie son lot de drames contre lesquels nous devons lutter. Au cours de l'examen de ce texte en première lecture, la majorité sénatoriale est revenue sur deux dispositions phares : la réécriture de la définition du viol et la suppression du caractère contraventionnel de l'outrage sexiste au profit du caractère délictuel.

Cet accord symbolise une volonté commune forte en faveur du renforcement de l'arsenal juridique et de la fixation d'interdits sociaux clairs dans la loi. À cet égard, je tiens à saluer le travail des rapporteurs des deux chambres, des députés et des sénateurs qui a permis, malgré les divergences initiales, d'aboutir à un texte équilibré. Tout d'abord, la réécriture de l'article 2 facilite la caractérisation de la contrainte morale et de la surprise lorsqu'un acte de pénétration est commis par un majeur sur un mineur. Par ailleurs, dans l'hypothèse où la qualification de viol serait contestée, le président de la cour d'assises devra systématiquement poser une question subsidiaire sur la qualification d'atteinte sexuelle. Ainsi, l'auteur d'une infraction sexuelle ne restera pas impuni. Nous nous réjouissons aussi du rétablissement du caractère contraventionnel de l'outrage sexiste. Les forces de police pourront verbaliser immédiatement des comportements facilement identifiables, qui n'ont rien de la drague ou du compliment, par une amende qui pourra aller de 90 à 750 euros. Cette nouvelle rédaction permet d'assurer une répression immédiate des comportements abusifs. L'actualité nous ramène au harcèlement de rue que subissent régulièrement les femmes dans notre pays. Vendredi dernier, Mme Marie Laguerre a été victime d'un homme qui a incontestablement porté atteinte à sa dignité avant de la violenter. Elle a porté plainte contre cet homme, dont les actes seront certainement punis, conformément au dispositif juridique actuel. Alors, à quoi bon créer une amende pour outrage sexiste, me direz-vous ? ? À apporter une réponse immédiate si l'agresseur est pris en flagrant délit. On ne peut plus considérer comme dérisoires ces faits, qui sont malheureusement trop courants. Je tiens aussi, madame la secrétaire d'État, à saluer l'avancée proposée par le Sénat qui fait de l'orientation sexuelle de la victime une circonstance aggravante de l'outrage sexiste. Je me félicite également des dispositions qui ont été conservées : l'allongement du délai de prescription de vingt à trente ans pour les crimes commis sur mineurs ; la création d'une circonstance aggravante lorsqu'une infraction sexuelle est commise sur une personne vulnérable en raison de sa situation économique ou lorsqu'elle a entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; la création d'une nouvelle circonstance aggravante lorsque les victimes d'infractions sexuelles se sont vu administrer des substances nuisant à leur intégrité physique ou psychique ; la création d'un délit de captation d'images impudiques pour sanctionner les personnes filmant les femmes à leur insu dans les transports en commun ou ailleurs. La définition du harcèlement sexuel a également été enrichie par la réintégration de la notion de propos sexistes, et nous nous en félicitons. Le texte final, fruit d'un accord transpartisan, jouera un rôle majeur pour une meilleure protection de nos enfants et contribuera à reconnaître et à réprimer le fléau qu'est le harcèlement de rue. Pour ces raisons, madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le groupe La République En Marche votera en faveur de ce texte. La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voici donc au terme d'un débat ô combien médiatique, dont nous avons été saisis plusieurs fois ces derniers mois : d'abord à l'occasion de l'examen de la proposition de loi de M. Bas, suite de la mission d'information conduite par Mme Mercier, puis par le Gouvernement, qui nous a présenté le mois dernier un projet de loi largement revu après l'avis du Conseil d'État. Réunie au Sénat lundi dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord, en reprenant largement les dispositions adoptées par la Haute Assemblée. Pour ce qui est du contenu du texte, nous sommes plutôt satisfaits, celui-ci ayant été, selon nous, amélioré par le Sénat. En effet, même si le texte final ne retient pas la promesse initiale du Gouvernement qui établissait un seuil de non-consentement à un acte sexuel pour les mineurs de moins de quinze il ne reprend pas non plus le très polémique délit d'atteinte sexuelle avec pénétration qui pouvait laisser craindre que l'on ne minore les faits de viol. Cette disposition a été supprimée dès la discussion générale au Sénat par Mme la secrétaire d'État. La commission des lois et la majorité sénatoriale ont cependant clarifié la définition du viol en ajoutant une notion de présomption de contrainte qui tient compte de la différence d'âge entre le mineur et le majeur, ainsi que de la vulnérabilité et du discernement du mineur. a été préférée à la création d'un crime de violence sexuelle sur enfant soutenue par la délégation aux droits des femmes du Sénat et plusieurs sénatrices du groupe CRCE. Si l'ensemble de mon groupe ne partageait pas forcément toutes les demandes des associations sur le sujet, en particulier l'aggravation des peines, nous sommes unanimes sur un point

le Gouvernement, comme la majorité des parlementaires, s'est employé à aggraver les peines en matière de délits et crimes sur mineurs, ne portant que très peu d'intérêt à la prévention et à l'éducation. Or le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, tout comme celui de la protection des mineurs, ne saurait être circonscrit au seul angle répressif. Les volets préventif et éducatif doivent être exploités bien davantage. Ils sont la clé du mieux vivre ensemble et de l'évolution des moeurs. nous nous félicitons de l'adoption de quelques-uns de nos amendements. Je pense en particulier à celui qui tendait à renforcer l'article L. 312-16 du code de l'éducation, lequel dispose que trois séances d'éducation à la sexualité doivent être dispensées chaque année dans les écoles, les collèges et les lycées. L'éducation à la sexualité constitue un levier de lutte contre les discriminations. Elle doit être non pas réduite aux seules dimensions physiques et biologiques, mais appréhendée de manière globale. L'éducation doit contribuer, dès le plus jeune âge, à détruire stéréotypes et préjugés, mais nous sommes aujourd'hui encore loin du compte. Aussi, s'il est besoin de légiférer, c'est selon nous essentiellement en ce sens. Toujours plus de répression ne réglera rien au fléau des violences faites aux femmes ou aux enfants si le problème n'est pas pris dans son ensemble. Or cela ne pourra prendre forme qu'avec la discussion d'un projet de loi-cadre sur le sujet, que nous soutenons depuis un certain nombre d'années avec les associations féministes, notamment le Conseil national pour le droit des femmes. Enfin, alors qu'une importante réforme de la justice sera discutée- en tout cas nous l'espérons -dès cet automne, j'alerte l'ensemble de nos concitoyens sur cette conception du droit pénal, qu'il s'agirait de modifier sans cesse au gré des faits divers pour aggraver les sanctions, sans tenir compte ni du sens

depuis maintenant un an, à l'échelon tant international que national, le tabou des violences sexuelles faites aux femmes est tombé, permettant une prise de conscience de l'ensemble de notre société. Cette prise de conscience est d'ailleurs remontée jusqu'au sommet de l'État, puisque le Président de la République a fait de ce combat une grande cause nationale du quinquennat. Je me réjouis que la CMP sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ait été conclusive. J'aimerais plus particulièrement souligner l'engagement de Mme la rapporteur, Marie Mercier, et du président Philippe Bas, qui avait déjà impulsé ce débat grâce à une proposition de loi adoptée par notre assemblée, à une large majorité, au début de l'année. Je souhaite également souligner le travail important engagé par la délégation aux droits des femmes, sous l'égide de sa présidente, Annick Billon, et, enfin, saluer votre implication, madame la secrétaire d'État, sur un sujet, qui, je le sais, vous tient à coeur. Quels sont, après cette commission mixte paritaire, les points importants à retenir ? À titre personnel, je regrette que la proposition faite par la délégation aux droits des femmes concernant la création d'un crime de pénétration sexuelle sur mineur de moins de treize ans par un adulte n'ait pas été retenue. De même, il est regrettable que l'inversion de la charge de la preuve, proposée par la commission des lois du Sénat, ait été rejetée. Le texte se limite, pour les mineurs de moins de quinze ans, à préciser que la contrainte et la surprise seront caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. C'est déjà ça ! Pour autant, il nous faudra continuer à travailler sur les questions de présomption et de consentement des mineurs dans le cadre des crimes sexuels, afin de parvenir à une protection totale de nos enfants, comme ont pu le faire certains de nos voisins européens.

En effet, nous le savons, les victimes ont besoin de temps pour saisir la justice en raison du traumatisme causé par ces agissements, d'autant plus lorsque les faits ont lieu durant l'enfance. De plus, toujours en matière de prescription, j'ai bien noté l'engagement pris par Mme la ministre de la justice de publier une circulaire pour que, sur l'ensemble du territoire, les procureurs puissent ouvrir une enquête, malgré la prescription des faits. Ce dispositif permettra de vérifier que l'auteur présumé n'a pas commis d'autres infractions sexuelles, qui, elles, ne seraient pas prescrites. Ainsi, ces actes ne resteraient pas impunis. Autre point important : l'abandon de la création d'un délit d'atteinte sexuelle avec pénétration qui risquait de favoriser la correctionnalisation des viols relevant normalement de la cour d'assises. En effet, ce point avait suscité une grande inquiétude chez les associations et les représentants des victimes, qui craignaient que ce dispositif ne soit utilisé à mauvais escient, rendant plus complexe la caractérisation d'un viol. Soulignons aussi la pénalisation de l'administration de substances afin d'altérer le discernement et le contrôle d'une personne, pratique malheureusement répandue chez les prédateurs sexuels, ou encore la prise en compte de la situation de détresse économique comme circonstance aggravante, introduite par notre collègue Laure Darcos.

Le texte permet également de définir un cadre juridique précis en matière de harcèlement sexuel et moral, en tenant compte, notamment, des nouvelles formes de violences numériques, qui, nous le savons, sont particulièrement répandues chez les plus jeunes. Relevons encore l'ajout des violences intrafamiliales en circonstance aggravante pour un certain nombre d'infractions, ainsi que la sensibilisation des enfants à ces violences, par le biais de l'éducation nationale, car il faut un lieu où l'on puisse apprendre que parfois, ce que font papa et maman à la maison n'est pas toujours une pratique normale. La création d'une infraction pour outrage sexiste afin de punir également les comportements que subissent les femmes quotidiennement, notamment les diverses formes de voyeurisme, est une avancée majeure. À partir de ce jour, il est illégal d'aller regarder sous les jupes des filles. Enfin, notons l'inscription dans la loi de la lutte contre les mutilations sexuelles, suivant les recommandations du rapport réalisé par Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac. Il est en effet intolérable qu'encore aujourd'hui une femme soit excisée toutes les quinze secondes dans le monde, et que cette pratique ait aussi lieu sur notre territoire. En conclusion, un regret, des satisfactions, mais vous l'aurez compris, le groupe Union Centriste votera le présent projet de loi.

nous étions interrogés sur l'ambition réelle du Président de la République concernant la lutte contre les violences faites aux femmes, mais surtout s'agissant de l'égalité entre les femmes et les hommes,

de l'outrage sexiste. Cette question a été remise dans l'actualité- j'ai envie de dire « tant mieux ! » pour ceux qui n'ont pas encore compris de quoi nous parlions -avec ce fait divers du week-end qui a permis à chacun de voir en vidéo ce qu'était le sort des femmes dans la rue lorsqu'elles s'avisaient

Ont été retenues, notamment, les propositions socialistes concernant le cyberharcèlement. En revanche, certaines dispositions, qui nous semblaient importantes, et qui avaient été adoptées par le Sénat, ont finalement été retirées. C'est, par exemple, le cas de l'obligation de signalement de mauvais traitements sur enfants,

Nous espérons que votre ambition incontestable, madame la secrétaire d'État, se concrétisera lors de textes à venir. Nous ne mettons pas en doute votre volonté de lutter contre des comportements

terminer, je veux saluer une instance du Sénat qui a fait un travail formidable. Je veux parler de la délégation aux droits des femmes, qui a, de façon transpartisane, comme notre groupe de travail de la commission des lois, contribué à sa manière, avec un succès inégal,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, le Président de la République a fait de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes une cause nationale- c'est un engagement fort et nécessaire de la République

protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles. Ces deux contributions furent le fruit d'un groupe de travail pluraliste, dont je tiens à saluer la qualité des réflexions.

mais également à la plupart des propositions issues du groupe de travail, telles que l'allongement à trente ans du délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs et le renforcement des peines encourues pour atteinte sexuelle. me félicite que de tels apports du Sénat aient été retenus. Concernant la lutte contre le cyberharcèlement plus précisément, l'article 3 adapte opportunément notre droit pénal aux évolutions technologiques, en complétant la définition du harcèlement pour prendre en compte les « raids numériques », c'est-à-dire la

que la lutte contre le cyberharcèlement constitue un véritable enjeu en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Ces agressions ne sont en rien virtuelles. Bien au contraire, elles se révèlent tout aussi graves que des violences physiques et présentent des spécificités qui les rendent encore plus nuisibles pour les comme la difficulté à identifier des agresseurs protégés par leur anonymat et le potentiel de diffusion élargi des contenus. la définition actuelle du harcèlement, qui suppose la répétition, ne permet pas de réprimer de tels agissements, puisque les auteurs des « raids » réitèrent rarement les mêmes propos, mais se coordonnent afin de cibler, de manière collective, la même personne.

contester la légitimité. Nous sommes tous convaincus, au sein de cet hémicycle, de la nécessité de donner un coup d'arrêt à un certain nombre de violences, confinant parfois à l'inhumain, et qui continuent à se produire. Qu'elles concernent les mineurs ou les majeurs, qu'elles se déroulent sur internet, au travail, en public ou dans la rue, toutes les violences sexuelles et sexistes doivent être dénoncées et combattues avec fermeté. Aussi, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants-République et

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, madame la rapporteur, vous l'avez rappelé, mes chers collègues, l'actualité nous a démontré l'importance des violences sexuelles et sexistes et plus précisément du harcèlement de rue. Si le témoignage de Marie, agressée pour avoir osé répondre à un comportement inqualifiable, doit nous révolter, nous inquiéter, il doit surtout nous alerter sur toutes ces femmes, victimes chaque jour de ces agressions et qui se taisent, par honte, par dégoût et, parfois même, par crainte de ne pas être prises au sérieux. À l'heure où 80 % des victimes des violences sexuelles sont des femmes, le projet de loi qui nous est présenté nous oblige à la gravité et nous conduit à réfléchir aux solutions à trouver pour mettre fin à ces agissements. des membres de cet hémicycle a partagé avec vous, madame la secrétaire d'État, le même objectif : mieux protéger les victimes et condamner plus fermement les auteurs d'infractions sexuelles et sexistes. Je me réjouis d'abord que nous soyons tombés d'accord sur l'allongement du délai de prescription de l'action publique pour les crimes et délits d'agressions sexuelles qui passe de vingt à trente ans. Cette mesure est, à mes yeux, la principale avancée de ce projet de loi, sûrement la plus significative. Il est aujourd'hui nécessaire de prendre en compte la difficulté que peuvent rencontrer les victimes à parler tout de suite, car nombre d'entre elles enfouissent leur traumatisme durant des années. regret concerne la suppression de la présomption de contrainte conduisant à qualifier une relation sexuelle de viol dans deux cas : lorsqu'il y a un manque de discernement de l'éventuelle victime et dans le cas d'une différence d'âge significative entre l'auteur majeur et le mineur.

1 A annexant au projet de loi le rapport sur les orientations de la politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Cette disposition que l'on devait à notre rapporteur, Marie Mercier, enrichie par la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des sens, davantage de corps et de profondeur au présent texte, notamment parce que le rapport posait un cadre pour la prévention et une meilleure prise en compte de l'accueil des victimes. Le choix qui a été fait de définir plus précisément les circonstances aggravantes, notamment par la prise en considération, comme le souhaitait le Sénat, de la différence d'âge significative

elle partait d'une bonne intention, laissait planer le risque de la correctionnalisation. À ce titre, nous ne devions prendre aucun risque. Quant à l'article 2 C, nous restons pleinement en phase avec les dispositions tendant à alourdir les peines en cas de non-assistance et de non-dénonciation des crimes et délits commis contre l'intégrité corporelle des mineurs de quinze ans. Ces mesures reprennent là aussi nos travaux réalisés en mars dernier. Une partie des membres de mon groupe regrette toutefois la suppression de l'obligation pour les médecins de signaler les violences sexuelles. Aujourd'hui encore, on sous-estime le rôle de ces derniers dans la dénonciation de ces infractions, alors même qu'ils sont des professionnels de confiance et des interlocuteurs privilégiés. S'agissant des dispositions relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral, je tiens à rappeler notre soutien aux mesures visant à condamner les raids numériques. Sera désormais réprimé le comportement de plusieurs individus harcelant de manière unique, mais collective, une victime. C'est, par exemple, souvent le cas sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter. la définition du harcèlement sexuel, si certains d'entre nous sont favorables à l'élargissement proposé par l'Assemblée nationale, d'autres continuent de craindre que cette extension ne vienne créer la confusion avec le délit d'outrage sexiste prévu par l'article 4.

Cette prévention est d'autant plus primordiale dans un contexte où la moitié des infractions sexuelles sur mineurs sont commises par des mineurs. Il faut également lutter de toutes nos forces contre la pédophilie et la pédopornographie. Si des initiatives existent à l'échelle mondiale- je pense à la base de données internationale sur l'exploitation sexuelle des enfants d'Interpol -, l'idée de créer une structure française de prévention et de lutte contre la pédophilie- elle a fait l'objet d'une question au gouvernement de ma collègue Françoise Laborde -mériterait d'être étudiée avec plus d'intérêt. le viol enfin, il faut insister sur l'accompagnement des victimes, et ce dès le départ, avec la généralisation des salles Mélanie, davantage de moyens et de publicité pour les associations spécialisées. Il faut également aller plus loin dans la libération de la parole ! Si le nombre de signalements est en augmentation, nous ne pouvons nous en réjouir. Ces chiffres nous donnent le nombre d'auteurs, mais ne nous informeront jamais sur le nombre de victimes, car, aujourd'hui encore, beaucoup d'entre elles se taisent. Vous l'aurez compris, il nous reste encore beaucoup à faire pour que cessent les violences sexuelles et sexistes. L'adoption de ce projet de loi, à la suite de la réussite de la commission mixte paritaire, doit être considérée non pas comme une fin, mais comme un moyen, une arme supplémentaire dans l'arsenal législatif pour lutter contre ces comportements.

la commission mixte paritaire. Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement

Le scrutin est ouvert.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

L'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie

ministre de l'intérieur, qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui en raison de sa présence à l'Assemblée nationale, aux côtés du Premier ministre, pour le débat sur les motions de censure. Chacun comprendra que sa présence à l'Assemblée nationale était indispensable. Après l'échec de la commission mixte paritaire, qui, le 4 juillet dernier, n'est pas parvenue à un accord, l'Assemblée nationale a examiné, en nouvelle lecture, le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Elle a adopté jeudi dernier une version rétablissant les grands équilibres auxquels elle était parvenue en avril dernier,

Conformément au dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, il appartient désormais au Sénat de se prononcer en nouvelle lecture dans des délais que je sais particulièrement contraints, mais qui découlent de la volonté du Gouvernement d'achever l'examen parlementaire de ce texte avant l'été, afin que les mesures qu'il contient puissent rapidement entrer en vigueur. Au cours de sa réunion de ce matin, votre commission des lois, tirant les conséquences de l'échec de la commission mixte paritaire, a décidé de proposer au Sénat l'adoption d'une motion tendant Le Gouvernement prend acte de cette décision et ne pourra que se plier à la décision que la Haute Assemblée rendra tout à l'heure. Je veux dire solennellement que le Gouvernement aurait largement préféré que les assemblées parviennent à un accord. que vous y avez travaillé dans le cadre d'un dialogue constructif avec les députés, la majorité de l'Assemblée nationale ayant notamment proposé un certain nombre de compromis. Toutefois, concernant certains grands choix politiques défendus par le Sénat, qu'il s'agisse de l'instauration de quotas ou du remplacement de l'aide médicale de l'État par une aide médicale d'urgence, le Gouvernement et sa majorité ne pouvaient y souscrire. Dès lors, face à une telle situation de blocage, la commission mixte paritaire n'a pu que tirer les conséquences de ces désaccords, nous le regrettons ... peut-être tous d'ailleurs Il est désormais temps d'avancer. Cela fait près d'un an que les grandes options retenues par le Gouvernement en matière d'asile et d'immigration font l'objet de débats, depuis la présentation par le Premier ministre, le 12 juillet 2017,

dans l'hébergement d'urgence et l'accueil des demandeurs d'asile. Le ministre d'État et moi-même avons, du reste, longuement consulté et écouté le milieu associatif au cours de cette période. Le projet de loi est, quant à lui, connu depuis le 21 février dernier, date de son passage en conseil des ministres. Il a fait l'objet de débats intenses et nourris en commission et en séance publique, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Il a été largement amendé, précisé et enrichi ; et je dois dire que la version qui vous est aujourd'hui soumise est le fruit des travaux parlementaires. Après le temps de la discussion parlementaire, le Gouvernement considère qu'il faut désormais passer au temps de l'action. Car s'il est un enjeu au coeur des préoccupations des Français sur lequel il est indispensable d'apporter des solutions, c'est bien celui de l'asile et de l'immigration.

à 600 000 personnes, il a cependant continué à augmenter en France, avec 100 000 demandeurs en 2017, ce qui représente une croissance de 17 % en un an. Les conséquences de cette évolution, les Français les vivent au quotidien parce que le parc d'hébergement des demandeurs d'asile est saturé, que celui de l'hébergement d'urgence l'est tout autant et que se développent dans le coeur de nos villes le coeur de nos villes des campements dont chacun sur ces travées s'accorde à dire qu'ils sont indignes de notre République. Pour faire face à cette situation de plus en plus intenable, le Président de la République et le Gouvernement interviennent sur tous les fronts. Nous agissons à l'échelon international pour contribuer à la stabilisation de la rive sud de la Méditerranée et pour faire en sorte, au travers de l'aide au développement, que la jeunesse des pays africains puisse trouver un avenir. En outre, par une coopération étroite avec les États africains, nous pourrons mieux lutter contre les filières de passeurs qui font trafic d'êtres humains. Nous agissons également au plan européen pour rapprocher les législations des États membres, pour consolider le régime d'asile

ne voient pas un certain nombre de leurs ressortissants détourner cette disposition en déposant des demandes d'asile abusives. Ces mesures sont indispensables, car c'est évidemment à l'échelon européen qu'il faut concevoir les réponses à apporter aux défis migratoires- chacun a pu voir à quel point la question migratoire était de nature à mettre profondément en question les relations entre les États au sein de l'Union européenne. aussi indispensable que nous revoyions nos propres politiques qui ne fonctionnent plus. La France doit continuer à être une terre d'accueil pour toutes celles et tous ceux qui fuient la guerre et les persécutions ; mais nous devons aussi éloigner de notre territoire celles et ceux qui n'ont pas de droit au séjour.

pourront commencer plus rapidement leur parcours d'intégration, tandis que ceux qui, au contraire, seront déboutés pourront regagner leur pays sans que les liens familiaux et sociaux avec leur pays d'origine se soient distendus. Réduire les délais d'instruction de la demande d'asile, c'est ce que vise ce projet de loi, et c'est aussi ce que nous avons commencé à réaliser dans les faits. Pour ne prendre qu'un exemple, le temps nécessaire pour obtenir un premier rendez-vous en préfecture est ainsi passé en quelques mois de vingt et un jours à moins de quatre jours seulement. les renforcements d'effectifs dans les services étrangers des préfectures, avec 150 équivalents temps plein, permettront de progresser encore sur cette voie. Il fallait aussi gagner en efficacité pour ce qui concerne nos politiques d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Vous le savez, grâce à la mobilisation des préfets et de l'ensemble des services, le nombre de personnes ayant quitté le territoire a augmenté de 21,6 % en un an. Enfin, dans le cadre de la loi de finances pour 2018, nous avons mobilisé les moyens budgétaires qui vont nous permettre à la fois d'héberger dans des conditions dignes les demandeurs d'asile d'asile et de mieux intégrer celles et ceux qui ont vocation à rester sur notre sol au travers, notamment, du renforcement des cours de Français. Nous en sommes persuadés, avec ce projet de loi, nous apportons la bonne réponse, une réponse qui ne nie pas les problèmes que nous connaissons en matière d'asile et d'immigration, mais entend leur apporter des solutions équilibrées. Nous avons largement débattu du contenu de ce texte. Aussi ne reviendrai-je pas en détail sur les différentes mesures que comporte celui-ci. Si l'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, rétabli en très grande partie les dispositions qu'elle avait adoptées le 22 avril dernier, elle a retenu plusieurs modifications du texte adoptées par le Sénat.

réfugiés et apatrides, de refuser ou de mettre fin au statut de réfugié en cas de condamnations pour des faits graves, notamment de terrorisme, prononcées dans un autre pays de l'Union européenne, que l'obligation pour l'Office de statuer en procédure accélérée quand le demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. l'article 5 qui consacre dans la loi les opérations de réinstallation dans les pays tiers, organisées par les autorités en charge de la politique de l'asile.

la mise en place d'une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de l'éducation nationale, de gestionnaires de lieux d'hébergement et d'associations de défense des droits des demandeurs d'asile, commission qui émettra un avis sur les schémas régionaux d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés. des articles 9 et 9 issus de la proposition de loi déposée par M. Thani Mohamed Soilihi, qui a pour objet d'adapter l'application du droit du sol à Mayotte, compte tenu de l'ampleur de l'enjeu migratoire dans l'archipel. Le Gouvernement étant très attentif à la situation mahoraise et déterminé à apporter des solutions pragmatiques à cette problématique migratoire spécifique, nous avons, dans le droit fil des propos tenus par le chef de l'État, décidé de soutenir ces dispositions. mentionner l'article 26 autorisant la constitution d'un traitement de données comprenant les empreintes digitales et la photographie des personnes se présentant comme des mineurs non accompagnés, dans le double objectif d'assurer la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers. Il me semblait important de rappeler ces apports voulus par le Sénat, qui a été entendu sur tous ces points. S'agissant du placement en rétention des familles accompagnées de mineurs, sujet délicat qui touche chacune et chacun d'entre nous, le Gouvernement a pris bonne note de la solution retenue par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Si votre Haute Assemblée avait décidé de limiter à cinq jours le placement en rétention des mineurs accompagnés de leurs parents, le Gouvernement avait fait valoir les difficultés opérationnelles qui pouvaient s'opposer à une telle limitation. Je crois d'ailleurs que celles-ci avaient été entendues.

à une procédure d'éloignement. Il est toutefois nécessaire de la prévoir, car c'est le seul moyen pour faire appliquer le droit Bien entendu, dans ces cas, nous veillerons à ce que celle-ci s'effectue dans des locaux adaptés, uniquement destinés à l'accueil des familles, et à ce qu'elle soit toujours la plus brève possible. le Gouvernement a entendu les préoccupations exprimées par les députés et les sénateurs et demeurera attentif, dans le cadre d'initiatives législatives qui pourraient intervenir prochainement, aux équilibres entre ces différentes exigences. Je veux, pour terminer, souligner que l'Assemblée nationale a rétabli l'article 19 du projet de loi relatif au prétendu « délit de solidarité », article qui avait été supprimé par le Sénat. Les députés étaient d'autant plus fondés à le faire qu'il était nécessaire de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet dernier. En effet, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions existantes, au motif que l'exemption pénale et du droit d'asile pour l'aide accordée aux personnes en situation irrégulière ne s'étendait pas à l'aide à la circulation. Il a rappelé bien sûr que cette exemption ne doit s'appliquer que si l'aide poursuit un but humanitaire. Or tel était précisément l'objet principal de l'article 19 voulu par les députés qui ont, de surcroît, adopté un amendement tire les conséquences de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel sur le fait que tout acte en relation avec une aide au séjour ou à la circulation, apportée dans un but humanitaire, ne saurait faire l'objet de poursuites pénales. Le Gouvernement relève enfin que la décision du Conseil constitutionnel rappelle bien que « l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle » et que, à ce titre, l'aide à l'entrée, et donc au franchissement de la frontière, doit demeurer pénalement répréhensible. Voilà ce que je souhaitais faire valoir en introduction de ce débat. Je relève que, malgré les points de convergence auxquels nous sommes parvenus, les désaccords entre le Gouvernement et la majorité sénatoriale, dont certains membres me semblent étrangers à l'efficacité des politiques publiques, ont prévalu. La parole

Aucun accord n'a pu être trouvé entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et le texte qui nous revient aujourd'hui est celui de l'Assemblée nationale. Je tiens à rappeler que, Je tiens à rappeler que, en première lecture, nous avions largement réécrit ce texte en élaborant, si ce n'est un contre-projet, en tout cas un nouveau projet qui nous paraissait plus cohérent, plus ferme et plus réaliste pour notre politique migratoire. Ce texte tendait notamment à renforcer les peines complémentaires d'interdiction du territoire, à réduire le nombre de visas accordés aux pays les moins coopératifs, qui font échec aux procédures d'éloignement de leurs ressortissants en refusant de délivrer les laissez-passer consulaires, à réintroduire la visite médicale des étudiants étrangers, afin de répondre à un grave enjeu de santé publique, à réorganiser la durée de la rétention administrative, interdire le placement en rétention des mineurs isolés et, enfin, à encadrer rigoureusement celui des mineurs accompagnant leur famille. La réduction de trente à quinze jours du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, prévue par le Gouvernement, mais que nous avons considérée comme étant attentatoire aux droits des demandeurs d'asile et inefficace, avait été supprimée. En outre, un effort particulier avait été consenti en faveur de l'intégration des étrangers en situation régulière, avec un investissement renforcé dans les cours de français et l'appui de Pôle emploi pour améliorer les dispositifs d'insertion sur le marché de l'emploi. Enfin, le Sénat avait souhaité soutenir et accompagner les collectivités territoriales en proposant l'insertion des places d'hébergement des demandeurs d'asile dans le décompte des logements sociaux prévu par la loi

La commission des lois du Sénat et moi-même regrettons que le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture ne prenne finalement que très marginalement en compte les préoccupations majeures exprimées par la Haute Assemblée. quelques points d'accord entre les deux chambres. Il faut insister sur le fait que l'Assemblée nationale a conservé le délai de trente jours pour interjeter appel des décisions de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile- c'est un point auquel nous étions attachés -, ainsi que l'adaptation du droit du sol à Mayotte. De même, il faut se féliciter de la création d'un fichier comportant les empreintes digitales et une photographie des étrangers se présentant comme des mineurs non accompagnés, même si cette initiative n'est pas tout à fait la même que celle que nous avions adoptée. Il n'en demeure pas moins qu'elle constitue une

J'ajoute que les désaccords entre l'Assemblée nationale et le Sénat sont malgré tout restés extrêmement nombreux. Le texte transmis aujourd'hui constitue une véritable occasion manquée- je le dis -en matière de lutte contre l'immigration irrégulière tout particulièrement il ne prévoit ni stratégie migratoire ni aucune des mesures de rigueur proposées par le Sénat. Je pense notamment à un meilleur encadrement de l'immigration familiale et à une plus grande efficacité des procédures dites « Dublin ».

De même, les politiques d'intégration demeurent le parent pauvre de ce texte, alors que l'Assemblée nationale aurait pu utilement s'inspirer des mesures de bon sens proposées par le Sénat, comme la certification du niveau de langue des étrangers

Des désaccords majeurs persistent également sur les modalités d'organisation de la rétention. Le séquençage adopté par l'Assemblée nationale à la fois peu protecteur pour les étrangers et trop contraignant pour l'autorité administrative et les tribunaux. Combien de fois nos services nous ont-ils

des mineurs accompagnants pourraient rester jusqu'à quatre-vingt-dix jours en rétention, puisqu'il s'agit du nouveau délai fixé par le texte. Nous avons également relevé un certain manque de considération pour l'action des collectivités territoriales en faveur de l'accueil des demandeurs d'asile,

la suppression du rôle de coordination des centres provisoires d'hébergement en matière d'intégration des réfugiés, et une mesure plus « exotique »- si vous me permettez cette expression à la tribune -, l'habilitation à légiférer par ordonnances pour réformer le contentieux des étrangers devant les juridictions administratives et créer des procédures d'urgence devant la CNDA.

de l'opposition, représentée ici par la majorité sénatoriale, n'ont pas été pris en compte, comme la transformation de l'aide médicale de l'État, le refus automatique du statut de réfugié en cas de motif d'ordre public, ou encore une disposition, en l'occurrence non normative, obligeant le Gouvernement à refuser des visas, alors qu'il s'agit d'une prérogative purement gouvernementale. Nous pouvons conclure que le dialogue entre les deux assemblées s'est déroulé positivement, normalement,

Éliane Assassi. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, alors que plusieurs mouvements populistes, voire néofascistes, creusent leur sillon au coeur de l'Europe, le dossier des migrants s'est installé ces derniers mois comme une thématique d'actualité importante et révélatrice d'une profonde crise au sein de l'Union européenne. Avec- certainement -en ligne de mire l'échéance électorale à venir et- justement -le scrutin européen de mai prochain, le Gouvernement et sa majorité En Marche défendent depuis avril un texte traitant à la fois du droit d'asile et du droit des étrangers, en s'attaquant aux droits fondamentaux et à la dignité humaine. Madame la ministre, je vous le dis d'emblée, les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste républicain citoyen et écologiste s'opposeront de nouveau très fermement à ce projet de loi, qui tend

sont réunies pour bafouer le droit d'asile et mettre à mal l'accueil de migrants à tout autre titre. Sans viser le même objectif précis, mais en tout cas en respectant les mêmes finalités générales, la majorité sénatoriale a fait adopter un certain nombre de mesures qui ont durci le texte et qui ont d'ailleurs fait échouer : l'introduction d'un vote parlementaire sur le nombre d'étrangers admis au séjour, par catégories, pour les trois ans à venir, la suppression de l'article 1 relatif à la délivrance de titres pluriannuels aux apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire, le durcissement des conditions de réunification et de regroupement familial, ou encore la suppression de l'aide médicale de l'État. Cependant, de l'économie générale du texte, il n'existe pas, selon nous, de profonde divergence entre les deux majorités parlementaires et, donc, entre la droite et le Gouvernement. Je rappelle que l'une des mesures les plus préoccupantes que le Sénat

au nom de l'unité du droit de la nationalité », ne fait que confirmer notre inquiétude ! Ainsi, l'équilibre revendiqué par la majorité à l'Assemblée nationale ne nous satisfait pas davantage et représente au contraire, pour nous, un leurre. Finalement, nous n'approuvons pas le texte, que ce soit dans sa version sénatoriale « aggravée

que nous avons effectuées. Aussi vais-je me borner à l'essentiel. La grande majorité de nos amendements a été rejetée : ils n'exprimaient pourtant pas une idée très révolutionnaire de notre politique migratoire. Il s'agissait simplement d'améliorer les conditions de vie et d'accueil des personnes, en respectant l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment aux droits fondamentaux : un toit, la santé, les besoins alimentaires ainsi que, éventuellement, les mêmes droits de recours que pour tout justiciable et un accès facilité au travail ... En outre, ces amendements veillaient à garantir le respect des principes fondamentaux auxquels notre pays a souscrit dans sa Constitution et dans ses engagements internationaux, considérant que, dans une Europe en proie à la montée des nationalismes, la France devait prendre ses responsabilités et réaffirmer les valeurs qu'elle a toujours défendues, et qui sont au fondement de notre République. Je le répète, car cela est suffisamment grave pour être répété autant que de besoin,

Une chose est sûre : ce projet de loi et les postures politiciennes adoptées par les uns et les autres ne proposent aucune issue à ce défi humanitaire et sont loin d'être à la hauteur. Croyez bien que nous le regrettons et continuerons à faire entendre notre voix en ce sens. Enfin, je finirai mon intervention par la seule bonne nouvelle de ces dernières semaines. Eh oui, il y a tout mon cher collègue ! Ah bon ? La fraternité devra désormais être respectée comme principe constitutionnel. Le Sénat s'honorerait à respecter la décision des sages en abrogeant totalement le délit de solidarité, qui n'est pas digne de notre devise républicaine. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères ! » écrivait Voltaire dans son. Mes chers collègues, face à l'obscurantisme de certains, puisse le siècle des Lumières continuer à nous éclairer

Notre analyse repose sur l'idée que l'échec des formations dites de gouvernement- ou de responsabilité -à trouver des accords sur ce type de sujet ne sert aucune d'entre elles, même quand elles sont dans l'opposition, et sert uniquement les extrêmes.

est, à notre sens, la tâche d'une génération et relève, donc, d'une logique qui doit être étudiée dans une perspective de long terme. Ce texte peine aussi à offrir une vision globale. Et pour cause ! Nous sommes devant des problèmes complexes, interdépendants, multifactoriels, avec des pays de départ, des pays de transit et des pays d'arrivée. La difficulté, pour l'exécutif comme pour le Parlement, est de travailler sur l'ensemble du dispositif

les accords entre États pour éviter les mouvements secondaires, l'hébergement, les délais d'accès, les délais d'instruction, la reconduction de ceux qui ne bénéficient pas du statut de réfugié et l'intégration de ceux qui en bénéficient. Oui, mes chers collègues,

Notre conviction est celle d'une souveraineté partagée. Il n'y a pas un volet communautaire, un volet intergouvernemental et, enfin, un volet franco-français. Pour nous, tout est lié. La souveraineté partagée sous-tend le renforcement de notre identité nationale comme de notre souveraineté d'État. Ce sont des éléments consubstantiels.

Parmi les problèmes que nous avons à traiter, la question des mouvements secondaires, souvent évoquée par notre rapporteur François-Noël Buffet, est très importante.

car les intéressés vont attendre, dans des conditions extrêmement négatives pour la société, l'expiration de ce délai pour faire une demande. Ce sont deux sujets sur lesquels, madame la ministre, nous vous demandons de vous faire notre interprète afin que les dispositifs

création de plateformes régionales de débarquement en dehors de l'Union européenne ou de centres dits « contrôlés » sur base volontaire au sein de l'Union européenne pour séparer les réfugiés considérés comme éligibles à la protection et les migrants économiques supposerait, bien sûr, de nouvelles dispositions législatives. Ce qui me semble important, madame la ministre, au risque d'insister une dernière fois, c'est que nous puissions avoir, sur cette problématique, non pas une vision technique- article par article, sujet par sujet -, mais une vision globale

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, voilà probablement l'un des sujets qui heurtent ou interrogent le plus notre responsabilité politique,

migrations. De tout temps, celles-ci ont favorisé l'activité économique, la connaissance et les échanges ! Dans la situation actuelle de la planète, il ne serait pas inutile de poursuivre une telle démarche ! Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi,

elle est prisonnière de ses peurs et complètement handicapée par celles-ci. Elle est affaiblie. Face à ses voisins et à ses partenaires, elle semble prête à renoncer

lutter à long terme contre l'immigration illégale sans accepter une certaine dose d'échanges intellectuels, familiaux, commerciaux, permettant de diminuer ces différences de potentiel qui, aujourd'hui, posent énormément de problèmes.

le retour de l'orientation directive sans hébergement garanti pour les demandeurs d'asile- une aberration absolue ! Comment peut-on obliger les gens à aller dans une région sans leur garantir d'hébergement

pas de prise en compte réelle et sérieuse du principe de fraternité rappelé par le Conseil constitutionnel ; acceptation de la compétence liée de l'OFPRA pour les remises en cause de statuts en cas de menace-

On remet en cause les principes du droit à la nationalité, qui s'appliquent à tous sur le territoire de la République,

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, éminemment sensible pour les Français, la question migratoire est devenue un enjeu de souveraineté nationale et de cohésion sociale. Illustration de cette importance, nos débats sur ces questions ont été longs, difficiles, passionnés, à la hauteur d'un enjeu fort pour nos concitoyens. Mais cet enjeu est également un enjeu pour l'Europe, nous avons eu l'occasion d'en débattre la semaine dernière à propos de l'accord de réadmission franco-autrichien. C'est l'avenir du « Vieux continent face à la jeune Afrique », comme je l'ai lu, qui est en jeu, un avenir qui ne doit pas verser dans la confrontation. L'Afrique subsaharienne compte déjà plus d'un milliard d'habitants, dont 70 % ont moins de trente ans. En 2100, trois bébés sur quatre qui viendront au monde naîtront au sud du Sahara. Comment, dans ces conditions, éviter une « ruée vers l'Europe », pour reprendre le titre de l'ouvrage récent de Stephen Smith, qui documente précisément cet enjeu ? Le vrai défi est là : réussir le développement d'un continent jeune et pauvre, séparé par un bras de mer d'un continent plus vieux et plus riche. Dans ces conditions, l'irénisme humanitaire me semble aussi dangereux que l'égoïsme national. Une approche équilibrée, globale et collective est nécessaire, sans verser dans l'outrance des parangons de vertu ou de ceux qui, comme dans la fable d'Ésope, crient tant au loup crient tant au loup qu'on ne les écoute plus. Cette nécessité de l'équilibre en matière de politique migratoire se retrouve dans une tradition républicaine, qui remonte au moins à la Libération. Depuis la signature de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par le général de Gaulle, il existe une continuité politique qui tente de concilier les impératifs proches, mais différents de la gestion de l'immigration, de l'intégration et du droit d'asile. En matière d'asile d'abord, la tradition républicaine repose sur une logique éthique que nous ne devons pas renier. Néanmoins, et c'est l'un des enjeux de ce texte, les procédures doivent être modernisées et les critères clarifiés pour éviter de laisser se développer des attentes infondées ou des situations indignes de notre pays. Je veux parler, par exemple, des conditions difficiles de travail à la Cour nationale du droit d'asile ou à l'OFPRA, des inefficacités de nos procédures de traitement et de la saturation de nos dispositifs d'hébergement, particulièrement en Île-de-France, dans les Alpes-Maritimes et dans le Pas-de-Calais. Quant à la question de l'intégration des étrangers dans notre pays, leur insertion linguistique, économique et sociale est particulièrement insuffisante en comparaison de certaines de certaines réussites chez nos partenaires, en Allemagne notamment. Dans un bel article de 1943 intitulé « Nous autres réfugiés », Hannah Arendt décrivait la situation la plus douloureuse pour le réfugié en terre d'accueil : l'exclusion, le rejet, l'anonymat. Et personne ici ne sait qui je suis ! », disait-elle. Nous devons faire en sorte que la promesse de l'accueil, une fois ses critères clarifiés, ne soit pas qu'une promesse procédurale ; qu'elle soit bien celle d'une insertion réelle. Nous avons déjà pu évoquer lors des précédents débats l'importance, dans ce cadre, du droit au travail. Sur le sujet de la maîtrise de l'immigration, le Sénat a proposé un texte qui est très éloigné de la version initiale du Gouvernement. Modifier ce texte n'était pas en soi une erreur, car on peut faire mieux que ce qui nous est proposé en matière d'exécution des décisions, de regroupement familial, de traitement des mineurs ou encore d'intégration. Je crois que nous sommes d'accord pour estimer que ce énième texte sur l'asile et l'immigration constitue un aménagement technique de notre droit qui ne résoudra pas la dimension structurelle du problème des migrations. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas important au contraire, il pourrait contribuer à changer en profondeur le quotidien des migrants et des agents de l'asile, dont l'engagement doit être salué. Sur ces questions particulièrement politiques, l'équilibre n'est pas simple à trouver entre, d'un côté, la nécessité d'humanisme, héritée de la tradition française des Lumières, qui demande d'accélérer les procédures et de moderniser le droit des étrangers et, de l'autre, la fermeté indispensable pour rendre les mesures d'éloignement plus réelles pour les déboutés. Tout au long de la discussion de ce projet de loi, nous avons souhaité conserver une approche mesurée, raisonnable. Nous voulons rappeler que la question migratoire doit être abordée en France, c'est l'objet de ce texte, mais aussi au niveau européen, sans lequel rien ne sera possible, et au sein des pays sources, tant le développement de ces derniers est une clef déterminante dans la résolution de ce sujet. Madame la ministre, mes chers collègues, nous devons en avoir conscience, la crise migratoire est encore devant nous, pour de nombreuses années. Et ce n'est qu'avec une réponse coordonnée à ces trois échelons que nous pourrons apporter une réponse empreinte d'humanité et de fermeté, lorsque cela est nécessaire, à la crise que nous connaissons.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la question migratoire est devenue l'une des principales variables des relations internationales.

est aujourd'hui instrumentalisée comme un puissant levier diplomatique par les pays bénéficiant de grandes diasporas ou stratégiquement placés sur les routes de l'exil. En Méditerranée, les flux migratoires conditionnent désormais les relations entre l'Union européenne et les pays du contour sud, à tel point que certains chercheurs, comme Henry Laurens et Manon-Nour Tannous considèrent que le pacte euro-méditerranéen n'est plus « qu'une triple mise à distance des États à qui l'on refuse l'adhésion, des migrants et des potentiels terroristes Cette importance croissante des migrations dans le monde nous impose de repenser en profondeur nos politiques étrangères de développement et de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi, et surtout, notre politique intérieure d'accueil et d'intégration des personnes étrangères, qu'elles sollicitent l'asile ou des titres de séjour de droit commun. Sur ce deuxième point, l'oeuvre de l'Union européenne est balbutiante, et l'on en constate tous les jours les limites. Dans nos centres de rétention administrative, les déficiences du système de Dublin sont encore plus palpables pour les agents chargés d'organiser les flux des reconduites à la frontière. À ceux qui sont exposés aux regards hagards et aux questions lancinantes d'individus perdus dans le labyrinthe administratif dublinois, comment expliquer les dysfonctionnements de procédures qu'ils ont pourtant la tâche d'exécuter ? Personne n'ignore ici l'impossibilité de rendre effectives toutes les reconduites à la frontière prononcées, tant que nos partenaires continueront de filtrer les retours par le biais des laissez-passer consulaires. Il est au demeurant peu probable qu'ils y renoncent, puisqu'ils manifestent ainsi leur souveraineté et le contrôle de leurs frontières. du RDSE, nous sommes comme vous attachés aux lois de la République, et nous sommes donc les partisans d'une exécution ferme des décisions administratives prises sur leur fondement. Ce que nous critiquions en première lecture, et ce que nous continuons de critiquer à ce stade des discussions, c'est la fragilisation de l'État de droit qui découlera nécessairement du renforcement des mesures dérogatoires figurant dans le texte issu des travaux de la commission des lois. Comme je le disais en première lecture, la dégradation des conditions d'accès à la justice des personnes étrangères les concerne en premier lieu, au mépris de leur incontestable vulnérabilité. Mais elle pourrait aussi menacer indirectement le justiciable français, si les expériences conduites en matière de droit des étrangers étaient généralisées devant nos juridictions. Nous craignons en particulier la généralisation du recours à la vidéo-audience, ce qui serait une transformation sans précédent du service public Fidèle à sa tradition, notre Haute Assemblée avait sur ce sujet introduit quelques dispositions protectrices utiles, comme l'encadrement du placement en rétention administrative des mineurs accompagnés et le rétablissement du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile à sa durée actuelle de trente jours. La navette a eu quelques vertus. Le maintien de cette deuxième disposition par nos collègues députés est une maigre consolation au regard des propositions de notre groupe et de nombreux collègues pour mieux protéger les enfants étrangers. Selon nous, le recours systématique à l'assignation à résidence était le meilleur compromis entre la protection de la minorité et la nécessité de mettre en oeuvre les procédures de reconduite à la frontière. Nous accueillons favorablement l'encadrement du « délit de solidarité », encore modifié par nos collègues députés en deuxième lecture, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel consacrant la valeur constitutionnelle du principe de fraternité. À ce stade, nous ne pouvons mesurer tous les effets contentieux que produira cette décision audacieuse, mais cela devrait nous conforter, en tant que membres du Parlement, dans l'idée qu'il ne faut pas renoncer au progrès des droits du citoyen en faisant preuve d'une autocensure excessive. Enfin, si l'atténuation brutale de l'afflux migratoire est peu probable et l'amélioration des reconduites aux frontières impossible, alors l'accueil et l'intégration deviennent incontournables. Ainsi, un usage plus constructif de l'aide au retour volontaire pourrait être fait, en ne l'appliquant qu'à moyen terme, afin de responsabiliser davantage les étrangers souhaitant rejoindre la France pour s'y former et y acquérir des compétences d'avenir. Cette relation de confiance, établie sur des règles claires, pourrait constituer le ciment d'un développement plus équilibré à travers le monde et favoriser un rayonnement singulier et positif de la France sur la scène internationale. Au contraire, ce projet de loi nous paraît complexifier un peu plus le droit des étrangers en France, et rester à la surface des enjeux migratoires. C'est pourquoi, comme lors de la première lecture, les membres du groupe du RDSE voteront contre ce texte, dans sa version modifiée par la commission des lois du Sénat.

que vous allez faire passer, madame la ministre, apparaisse complètement décalée par rapport à ce que certains États européens vont demander ou demandent déjà.

le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture n'a pris que très marginalement en compte les préoccupations majeures qui avaient été exprimées par la Haute Assemblée, ... Oui ! ... comme l'a d'ailleurs reconnu- j'allais dire presque loyalement -notre collègue rapporteur, Élise Fajgeles, à l'Assemblée nationale. À l'exception de l'accord trouvé sur le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le fameux délai d'un mois, et l'adaptation du droit du sol à Mayotte,

En deuxième lieu, le projet de loi constituait une véritable occasion pour lutter contre l'immigration irrégulière, et nous regrettons que cette opportunité n'ait pas été saisie.

De même, les politiques d'intégration demeurent le parent pauvre de ce texte, alors que l'Assemblée nationale aurait pu utilement reprendre des mesures que nous avions proposées,

Là, c'est tout à fait différent : il y a un texte issu de l'Assemblée nationale qui, si nous ne faisons rien, sera demain la loi.

Mes chers collègues, je suis en désaccord avec la façon dont nous fonctionnons par rapport à des textes comme celui-là. La procédure accélérée

dire. Pourquoi cette volonté constante de précipitation ? Il faut réformer ! Mon cher François Patriat, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je me souviens d'une période, pas si lointaine, où, dans cette assemblée,

est assez dramatique eu égard à la conception que nous avons du débat parlementaire. Je me souviens de dernières lectures où, conformément à ce qui est écrit dans la Constitution,

Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Personne ne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

la commission des lois a émis un avis favorable- 12 voix pour, 1 bulletin blanc -à la nomination de M. Jean-Raphaël Alventosa aux fonctions de médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques. mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire. M. le président du Sénat prendra acte de la clôture de cette session lorsque nous aurons reçu le décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement. Cette information sera publiée au et sur le site internet de notre assemblée. Sous réserve de la publication du décret de M. le Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire et de la communication de la lettre d'ordre du jour du Gouvernement,

Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous trente : Questions d'actualité au Gouvernement. À dix-sept heures quarante-cinq et le soir : sous réserve de sa transmission, suite de la nouvelle lecture du projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine,